d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous avons le plaisir d’accueillir dans notre tribune d’honneur une délégation de l’Assemblée nationale du Québec, conduite par sa présidente Mme Nathalie Roy.

La délégation est composée de M. Luc Provençal, vice président du groupe d’amitié, et de Mme Brigitte Garceau, tous deux députés. Elle est accompagnée par notre collègue Rémy Pointereau, le très actif président du groupe interparlementaire d’amitié France Québec. J’ai eu le plaisir d’échanger ce matin avec nos amis québécois, qui ont visité hier la Cité internationale de la langue française à Villers Cotterêts.

Mes chers collègues, en votre nom à tous, dans cette langue que nous avons en partage, permettez moi d’adresser un salut chaleureux à nos collègues de l’Assemblée nationale du Québec et de leur souhaiter un fructueux séjour

fonction publiques. Monsieur le ministre, l’inauguration, le 26 mars dernier, des locaux de l’agence de conseil interne de l’État pourrait être une bonne nouvelle. Je rappelle que, dans une anarchie déontologique absolue et une opacité complète, l’utilisation de cabinets de conseil avait coûté au contribuable plus de 1 milliard d’euros en 2021.

à l’Assemblée nationale – à reculons, il faut le dire, et bien détricotée… Pourquoi cette initiative en cours de navette parlementaire, alors que nous sommes en pleine disette budgétaire, que les agences et autres autorités pullulent à grands frais et que notre administration est dotée de nombreuses inspections générales, par ailleurs très compétentes ? Monsieur le ministre, en quoi cette agence interne va t elle régler les questions de transparence et éviter les consanguinités et les conflits d’intérêts ? Comment pourra t elle assurer une meilleure utilisation de nos ressources financières et des moyens de notre haute fonction publique ? La parole

Élaborer un plan de réinternalisation pour mieux valoriser les compétences internes et moins recourir aux cabinets de conseil. » Madame la sénatrice, c’est exactement précisément ce que nous faisons. À la vérité, nous pourrions nous rejoindre sur les objectifs. J’ai toujours été clair et constant sur ce sujet : il faut renforcer l’État et mieux maîtriser nos dépenses de conseil. C’est ce que nous faisons méticuleusement.

Monsieur le président, madame la ministre de l’éducation nationale, mes chers collègues, 1 500 ans : un établissement privé est susceptible d’être contrôlé une fois tous les 1 500 ans ! Oh, ça va ! Les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le contrôle des établissements privés sont sans appel. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur le double discours de votre gouvernement. D’un côté, vous donnez 7,8 milliards d’euros par an, sans aucun contrôle, à l’enseignement privé. De l’autre, vous rabotez le budget de l’école publique de 690 millions d’euros. Madame la ministre, quel est l’avenir de notre République sans l’école publique ? Chaque enfant doit recevoir des pouvoirs publics les mêmes moyens consacrés à son éducation et à son émancipation, quelles que soient son origine, sa position géographique ou ses croyances. Dans de nombreux territoires, l’éducation nationale n’est plus en mesure de garantir cette égalité des chances. En Seine Saint Denis, par exemple, le personnel éducatif, les parents et les élèves sont mobilisés depuis plus d’un mois. Leur demande est claire : ils souhaitent un plan d’urgence pour recruter et rénover les établissements insalubres. Votre réforme du « choc des savoirs » est un nouvel affront aux valeurs républicaines. En créant des groupes de niveau, vous institutionnalisez le tri social. Les conservateurs se sont toujours prévalus de la liberté d’enseignement pour s’opposer à la mixité sociale. Ils ont toujours agité le chiffon rouge d’une guerre scolaire. Aujourd’hui, ils usent de tous les artifices pour éviter le débat sur les ghettos scolaires. l’école de la République doit être un rempart face aux inégalités. Nous ne voulons ni des groupes de niveau ni de l’uniforme. Nous avons besoin d’un choc d’égalité et d’un choc de moyens. Nous attendons un plan d’urgence pour l’éducation nationale. Madame la ministre, allez vous remettre l’école publique au cœur des priorités de votre gouvernement ? Il faut conclure ! Dans quel camp êtes vous ? Celui des conservateurs ou celui des progressistes ?

Dans la diversité des mesures qui sont adoptées, il nous permettra, avec assurance, de prendre en charge la singularité de chacun de nos élèves, pour le porter au plus haut de ses compétences et de ses connaissances. Je le réaffirme devant vous. Par ailleurs, vous n’avez pas posé la question de la sécurité,

l’année dernière ? Au mois de novembre, pour être précise, les partenaires sociaux ont reçu une lettre de cadrage rédigée par le Gouvernement. Ce document a été préparé dans le contexte

quelque 3 millions d’emplois ont été créés et nous avons redoublé d’efforts pour réindustrialiser la France. Bref, tout va bien ! Certains reprochent au Gouvernement d’annoncer une nouvelle réforme de l’assurance chômage

C’est l’un des objectifs annoncés pour la réforme à venir, qui s’inscrit dans la poursuite des engagements du Gouvernement à bâtir un modèle social juste, où le travail paie toujours mieux que l’inactivité. Je tiens par ailleurs à rappeler aux commentateurs qui se focalisent sur la durée d’indemnisation que celle ci n’est que l’un des leviers envisagés dans les discussions en cours avec les partenaires sociaux. Il serait bon de laisser ceux ci travailler… En cristallisant le débat sur un seul paramètre, nous risquons d’occulter l’essentiel. Nous faisons confiance au dialogue social et nous saurons le retranscrire dans la loi, comme nous l’avons fait avec le consensus trouvé sur l’accord national interprofessionnel d’avril 2022. Espérons que les partenaires trouvent un accord pour dégager des solutions, afin que les Françaises et les Français au chômage puissent retrouver le plus rapidement possible le chemin de l’emploi madame la ministre, face aux critiques de cette réforme, pourriez vous nous préciser ses contours et nous indiquer comment elle aidera à atteindre l’objectif d’une société du plein emploi ?

Cela fait maintenant cinquante ans que l’État présente des budgets en déficit. Les collectivités territoriales, elles, les votent en équilibre. C’est la loi ! Pourtant, lundi prochain, le président du conseil départemental de l’Aisne proposera un budget en déséquilibre. Comme tous les départements, nous sommes affectés par la conjoncture économique. Mais, comme un certain nombre d’entre eux, nous sommes confrontés à des difficultés structurelles. Nous bouclons les budgets, ici, grâce à quelques millions d’euros issus des péréquations, là, avec quelques fonds de soutien exceptionnels… Cette situation n’est plus tenable. Depuis vingt ans, vous le savez, les départements assument en lieu et place de l’État une partie des politiques sociales et de l’accompagnement des plus vulnérables. Nous décalons les investissements dans les collèges. Nous ne pouvons pas consacrer les moyens suffisants aux routes. J’ajoute que, dans les départements ruraux, les collectivités locales doivent se substituer à l’investissement privé pour le déploiement de la fibre optique, pour racheter et maintenir le dernier commerce et pour investir dans la création de maisons médicales. médicales. Si l’on ne change pas le cadre, si l’on n’instaure pas une meilleure répartition des capacités à agir, si l’on ne fait pas régner une plus grande équité, si l’on ne remet pas le modèle à plat, un certain nombre de départements n’auront plus de raison d’exister et se contenteront d’être de simples de simples guichets sociaux. Monsieur le ministre, vous n’avez pas devant vous des élus qui viennent se plaindre de leur sort. Vous n’avez pas des gens qui sont dans une démarche politicienne, mais des responsables qui veulent une discussion utile pour bâtir des solutions pérennes. D’ailleurs, nous participons activement aux travaux de la mission Woerth. Monsieur le ministre, quelle réponse le Gouvernement compte t il apporter à ces départements qui sont au bord du précipice ? La

La diminution de leurs recettes, liée à l’effondrement des droits de mutation à titre onéreux, se conjugue à l’augmentation des dépenses sociales. Il y a des disparités entre les départements,

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le secrétaire d’État chargé de la mer, le 13 octobre 2017, nous assistions à la mise à l’eau de la première éolienne flottante en France, à Saint Nazaire, en Loire Atlantique. C’est une filière d’avenir. J’y crois et je veux que nous soyons l’un des leaders. » Tels sont les mots qu’a prononcés le Président de la République lors des dernières assises de la Mer, le mardi 28 novembre dernier à Nantes. Nous pouvons être fiers de posséder aujourd’hui en France les savoir faire et les entreprises susceptibles de construire les turbines, les pales et les sous stations nécessaires à l’atteinte des objectifs l’horizon n’est pas dégagé pour les acteurs de l’éolien en mer. Selon les grands industriels installés dans mon département, il y a un manque de planification et de visibilité pour atteindre l’objectif de 45 gigawatts en 2050.

en sont une parfaite illustration. Ayons bien en tête la situation catastrophique que connaît en ce moment la filière photovoltaïque en France : elle risque tout simplement de disparaître. Deux usines vont fermer dans mon département. Quelles sont les les mesures envisagées par le Gouvernement pour garantir une meilleure planification ? Plus précisément, concernant les appels d’offres, que prévoyez vous pour renforcer la compétitivité de nos entreprises face à la concurrence étrangère, notamment chinoise s’agissant de General Electric, que prévoyez vous pour accompagner ce creux de charge et permettre de conserver les 600 emplois et les savoir faire ? Enfin, monsieur le secrétaire d’État, vous êtes Breton comme moi. Vous êtes attaché à nos pêcheurs. Comment comptez vous rattraper les couacs de communication qui ont accompagné la présentation des cartographies des futurs parcs éoliens en mer ? Allez vous engager une véritable concertation avec les principaux acteurs concernés, en premier lieu avec les pêcheurs ?

– mener à bien ce travail de planification et lui donner de la visibilité. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer un méga appel d’offres sur l’éolien offshore de 10 gigawatts au mois de janvier 2025,

Lurel. Je dispose de deux minutes pour parler d’Haïti, un pays auquel notre histoire nous lie intimement depuis 1804, et des Haïtiens, qui, comme le rappelait Alexandre Dumas, n’ont cessé d’être Français qu’après avoir fourni leur « contingent de gloire » à la France. Haïti, vous le savez, est aujourd’hui au centre d’un cataclysme. Car quel pays pourrait résister à l’assassinat de son président, Jovenel Moïse, à une Assemblée nationale vide depuis 2023 et à la démission du septième premier ministre en l’espace de quatre ans le 11 mars dernier ? C’est un fait : le pays n’est plus dirigé. La mise en place d’un conseil de transition pour restaurer l’ordre public et démocratique dans un pays qui n’a pas voté depuis 2016, ainsi que de l’état d’urgence – il s’achève officiellement aujourd’hui

La République dominicaine, qui a déjà accueilli 700 000 Haïtiens et qui essaie d’endiguer l’afflux massif de réfugiés, mérite tout notre soutien. Face à la crise humanitaire, dont nous semblons avoir pris conscience tardivement, qu’attendons nous pour répondre à l’appel des Nations unies pour le déploiement d’une force internationale, à la fois pour protéger la population et pour créer les conditions d’une reprise du processus démocratique ? Six pays ont déjà proposé leur aide. Qu’entendez vous faire, madame la secrétaire

vous avez raison de souligner à quel point la situation sécuritaire en Haïti s’est fortement dégradée ces dernières semaines, avec des conséquences humanitaires catastrophiques. d’abord, je veux vous dire que la France condamne avec la plus grande fermeté les attaques des groupes criminels. Rétablir l’accès humanitaire est une priorité pour notre pays et pour l’Union européenne.

dans la constitution du conseil présidentiel de transition issu de l’accord de Kingston. Elle appelle désormais les membres du conseil présidentiel à désigner rapidement un nouveau Premier ministre pour établir la sécurité publique et préparer la tenue des élections.

ligne dans la lutte contre les groupes armés. La France a organisé à la fin du mois de mars dernier des affrètements spéciaux pour permettre aux ressortissants les plus vulnérables de quitter le pays. 243 personnes ont été prises en charge, dont 79 ressortissants étrangers. L’ambassade de France à Port au Prince continue de fonctionner et demeure pleinement mobilisée, au soutien de la communauté française sur place.

j’aurais aimé entendre un engagement de la France bien plus fort, en réponse à l’appel des Nations unies. Convenez en, la situation est intenable et ma question demeure sans réponse.

vous avez annoncé une nouvelle réforme de l’assurance chômage, la quatrième depuis qu’Emmanuel Macron a été élu, en 2017. Face aux déficits, vous cherchez 50 milliards d’euros. Et, plutôt que de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de taxer les super profits, vous cherchez encore une fois à faire des économies sur le dos des pauvres. Non, monsieur le Premier ministre, envisager une réduction de la durée et du niveau d’indemnisation, ce n’est pas inciter les gens à reprendre le travail ! Le chômage n’est ni un choix ni un confort. Il est toujours le résultat d’un accident de vie. Éloignement des bassins d’emploi, saturation du marché du travail et discrimination à l’embauche sont autant de problématiques qu’il faut régler en priorité. Le chômage ne s’explique pas par un prétendu attrait pour l’assurance chômage. Les chômeurs connaissent en réalité une double peine : celle des sentiments d’exclusion et d’inutilité et celle de la précarité. Ainsi, 35 % des chômeurs sont touchés par la pauvreté : ceux là sont deux à quatre fois plus nombreux en outre mer celles ci sont aussi des mères à la tête d’une famille monoparentale et, bien souvent, sans solution de garde, que vous allez, en contradiction totale avec les recommandations de la délégation aux droits des femmes, encore précariser. Dans un contexte d’inflation, de cherté de la vie et de crise du logement, les ménages les plus modestes doivent chaque jour choisir entre se loger et se nourrir. Appauvrir ces Français précaires, c’est créer encore plus de dettes locatives et d’expulsions. Comme l’a rappelé la secrétaire générale de la CFDT, le régime d’assurance chômage ne saurait être une variable d’ajustement budgétaire. J’ajoute que les chômeurs ne sont responsables ni du déficit ni de votre incapacité à gérer le budget de l’État.

Votre groupe n’était pas représenté à cet échange. La politique de la chaise vide ! Je reste ouvert à la discussion, pour que nous continuions à construire ensemble les économies nécessaires pour redresser nos finances publiques. Pas brillant Je vous ai bien écouté, monsieur le ministre, et je n’ai pas entendu de solution dans vos propos. Réduire le train de vie de l’État ? Oui, mais sur quoi ? Nous savons très bien que l’essentiel, c’est la masse salariale.

C’est cela, madame la ministre, les choix politiques et le projet de vie pour les Français de ce gouvernement : tout contre les assurés sociaux, tout contre les salariés et tout contre les plus pauvres, au bénéfice de ceux qui gagnent le plus et à qui l’on ne demande rien ! Les salariés s’en souviendront

M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. En ce cinquième anniversaire de la mort de Georges Pompidou, Président de la République auvergnat, sa réflexion est encore plus d’actualité : « Arrêtez d’emmerder les Français ! » Cinquante ans après, vous imposez à la ruralité le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement et le zéro artificialisation nette (ZAN) sur l’ensemble des territoires. Vous modifiez les zonages et les critères des zones de revitalisation rurale (ZRR). Monsieur le ministre, quelle écoute et quelle confiance accordez vous aux élus de nos territoires ruraux ?

dans la réalité, vous ne faites pas confiance aux élus. C’est toujours le « en même temps ». En ce qui concerne le ZAN, vous ne voulez céder en rien. Le Sénat vous propose la garantie rurale d’un hectare,

Vous vous enfermez dans ces certitudes d’une écologie punitive, muselant les élus des collectivités, qui n’auront plus la gestion de l’eau ni de l’urbanisme. En ne les écoutant pas,

Or il a été réformé en même temps que le a été supprimé. C’est cette année que la réforme entre en vigueur : l’épreuve écrite de fin de sixième année est remplacée par un concours écrit organisé en début d’année et un concours oral en fin d’année appelé Examen clinique objectif et structuré (Ecos). Cet examen oral consiste en une série de jeux de rôle, l’étudiant devant visiter des stations où l’attendent des patients interprétés par des volontaires rémunérés. L’intention est bonne, puisqu’il s’agit d’évaluer sa capacité à avoir les bons réflexes en situation. Malheureusement, les premiers Ecos blancs, organisés le 12 mars dernier, ont révélé de nombreux dysfonctionnements : étudiants interrogés par des connaissances ou même par des proches ; étudiants ayant trouvé le brouillon de leurs prédécesseurs d’une station à l’autre étudiants ayant entendu le passage des précédents au travers des cloisons ou de simples paravents ; fuite de sujets ; perte de grilles d’évaluation ; examinateurs ne connaissant pas leur rôle ou diffusant des indices… Bref, les défaillances sont nombreuses, et c’est une catastrophe qui rompt manifestement l’égalité des chances entre candidats. Dans ces conditions, quelles mesures comptez vous prendre pour que le concours de fin de sixième année, certainement le plus décisif de leur vie, où un centième de point peut faire la différence, ne s’apparente pas à une loterie ? À deux mois des examens seulement, une solution pourrait consister à rendre les Ecos validants, mais pas classants. Pourriez vous l’envisager ?

Madame la sénatrice Anne Sophie Romagny, vous avez raison de rappeler que ces épreuves sont une innovation dans le parcours de formation des futurs médecins.

L’examen blanc que vous avez mentionné était un test grandeur nature. Il a permis de déceler un certain nombre de dysfonctionnements – appelons un chat un chat – et d’envisager un certain nombre d’ajustements pour les épreuves qui auront lieu les 28 et 29 mai prochain.

Madame la ministre, les événements survenus au lycée Maurice Ravel de Paris, qui ont conduit à la démission de son proviseur, sont devenus le nouveau symbole de la lâcheté face à l’offensive islamiste. Le rectorat de Paris a maladroitement justifié son départ pour convenance personnelle, mais plus personne n’est dupe : ce proviseur a démissionné pour protéger sa sécurité, parce qu’il était la cible de menaces de mort et parce que, en 2020, un professeur, Samuel Paty, a été décapité,

Elle est bien plus que cela, car elle préfigure notre civilisation. Quand on défend la laïcité telle que notre République l’a conçue, on défend la cohésion nationale, le développement de l’esprit critique, les libertés individuelles et l’État de droit. Sur tous ces tableaux, si l’école sombre, c’est la France qui sombre.

le devoir de protection sociale et de solidarité est inscrit dans le préambule de notre Constitution ; ce n’est pas rien. On dit souvent que le degré d’une civilisation et d’une société se mesure à la manière dont y sont traités les citoyens les plus vulnérables ; j’ajouterai : ainsi que tous ceux qui les accompagnent. 1,3 million de travailleurs sociaux, dont 90 % de femmes, œuvrent au quotidien. Que leur dites vous ? Chacun de nous a été ou sera en contact avec eux ; chacun de nous aura besoin d’eux. Depuis des années, ces hussards bleus, blancs ou rouges de la République et de la solidarité alertent : le point de rupture est proche. Demain encore, ils manifesteront partout en France. Plus que de gratitude, ils ont besoin d’actes. Que leur direz vous ? La logique gestionnaire et les politiques de destruction sociale les fragilisent. Il est essentiel de mieux les rémunérer, de mieux reconnaître leurs compétences et de mieux les former. Que leur direz vous ?

sont dévaluées. Pour la première fois, des magistrats ont alerté sur la situation préoccupante du secteur de l’enfance. Devant le risque imminent de craquage du service social, quand présenterez vous enfin une feuille de route ambitieuse et budgétée pour retrouver la confiance de ces professionnels et tracer des perspectives ? Comptez vous intégrer au Ségur celles et ceux que vous continuez d’en exclure pour permettre une revalorisation salariale ? Enfin, en matière de protection de l’enfance, quand le décret établissant les taux et normes d’encadrement des établissements, prévu par la loi de 2022, sera

Les Républicains. Monsieur le ministre, je veux commencer mon intervention en saluant les nombreuses associations et institutions, ainsi que les départements qui œuvrent au quotidien pour une prise en charge de qualité des personnes handicapées. Malheureusement, en raison de la complexité administrative et de moyens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, ils ne peuvent apporter toutes les réponses. J’en veux pour preuve les articles ou les reportages mettant en exergue les problèmes que posent certaines conditions d’hébergement, de traitement et de soins dans le secteur du handicap. qui a été diffusé le 24 mars dernier sur M6 n’a laissé personne insensible. Quel choc ! Quelle indignité et surtout quelle honte ! Des enfants maltraités, des adultes malmenés, des parents interdits de visite, des conditions d’hébergement déplorables… Où en est la prise en charge des personnes handicapées ? Les mots ne sont pas assez forts pour dénoncer les nombreux dysfonctionnements d’un système qui laisse à l’abandon des personnes vulnérables, alors que celles ci, au contraire, devraient être une priorité dans notre pays.

personnes doivent être au cœur des actions à mener, il ne faut pas oublier leurs familles, qui, en plus d’être désemparées, sont bien souvent livrées à elles mêmes faute de place. Enfin, à l’heure où l’on parle d’inclusion, force est de reconnaître que celle ci n’est pas au rendez vous. Les témoignages de parents d’enfants autistes, notamment, en attestent. Face à ces difficultés, nous attendons des réponses. La ministre Fadila Khattabi a annoncé que tous les établissements sociaux et médico sociaux accueillant des personnes handicapées seront contrôlés que la parole des victimes sera libérée, et ce à partir de 2025. Désormais, nous attendons des garanties et des moyens. La

la seconde proposition de loi, vous la connaissez mieux que quiconque, puisque vous en êtes l’auteur. Au Sénat, nous avons introduit la possibilité de mener une expérimentation à l’échelle nationale

2024. Ah ! Pour répondre précisément à votre question, le décret élargissant la possibilité pour les infirmières de réaliser des certificats de décès à partir de l’expérimentation menée l’année dernière sera pris dans les prochains jours.

Le 27 mars dernier, nous apprenions la démission du proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel, dans le XX arrondissement de Paris. Le rectorat a indiqué qu’il s’agissait d’un simple départ en retraite anticipée pour convenance personnelle ; en réalité, il s’agissait d’une démission pour raison de sécurité. Ce proviseur avait reçu une multitude de menaces de mort après avoir demandé à une élève, le 28 février dernier, de retirer le voile qu’elle portait au sein de l’établissement. Cette dernière avait même prétendu que le proviseur l’avait violentée, et elle avait porté plainte. Tout cela était faux,

jours plus tard, donc, le proviseur démissionnait. Nous connaissons cette fabrique du mensonge. C’est exactement la même qui avait conduit à l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, et le CCIF était déjà impliqué. Jean Pierre Obin, auteur du fameux rapport, a déclaré qu’il s’agissait là d’une « victoire » pour les islamistes et d’un « épisode peu glorieux » pour la République. Depuis cette triste affaire, les messageries de centaines de lycées ont été noyées sous des menaces de terrorisme islamiste, et pas un jour ne se passe sans que de nouvelles menaces de mort envers la communauté éducative soient révélées. Elles ne représentent la partie émergée de l’iceberg, d’après un rapport sénatorial d’information paru voilà moins d’un mois. Par ailleurs, Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel, a récemment dénoncé le peu de progrès réalisés depuis ce qui est arrivé à son frère ; elle a mis en cause la responsabilité de l’État. Aussi, madame la ministre, ma question est simple comment comptez vous protéger les hussards noirs de la République face à l’entrisme islamique ?

intransigeants vis à vis des atteintes à la sécurité de notre communauté éducative. Je le redis devant vous : nos enseignants ne sont pas seuls. Nous sommes à leurs côtés,

pour l’ensemble des établissements. Ces actions structurantes s’articulent autour de trois axes. Premièrement, ce sont des actions de prévention. Pour cela, nous déployons évidemment des protections matérielles. Je le fais avec mes homologues des ministères de l’intérieur

en classe et en dehors de la classe. Bref, l’ensemble de ces dispositifs montrent que nous constituons un véritable bouclier auprès de nos équipes éducatives. Les enseignants ne sont pas seuls : nous sommes en permanence à leurs côtés. Madame la ministre, cela fait sept ans que le Gouvernement auquel vous appartenez est en charge de l’école et de la France, sept ans durant lesquels nous avons eu Samuel Paty, Dominique Bernard et de nombreux rapports qui n’ont jamais été suivis d’effet. Le 18 octobre 2020, le Président de la République Emmanuel Macron déclarait que la peur allait « changer de camp ». Rarement une prédiction aura été aussi peu aussi peu suivie d’effet… Dans ce domaine là comme dans tant d’autres, le constat de votre politique est celui d’un échec flagrant.

Acte est donné de votre mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion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 L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

la commission mixte paritaire (CMP) chargée d’élaborer un texte sur la proposition de loi de notre collègue députée du Morbihan visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels s’est réunie la semaine dernière et est parvenue à un accord, ce dont nous nous réjouissons. Ancré dans le quotidien de nos concitoyens, constituant souvent un irritant pour les élus et les chefs d’entreprise, le régime juridique de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage était jusqu’à présent de nature exclusivement jurisprudentielle.

permettra notamment d’exonérer de leur responsabilité des exploitants qui ont modifié leur activité de façon non substantielle ou pour se mettre en conformité avec les lois et règlements. Je ne puis m’empêcher, mes chers collègues, de vous raconter ce qui est arrivé dans mon département d’Ille et Vilaine,

à une rédaction qui, tout en visant des actes juridiques, demeure aussi large que possible. En contrepartie, nous avons fait droit à la demande d’un élargissement de la cause exonératoire prévue par le texte à l’ensemble des activités, et non plus aux seules activités agricoles.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, le texte dont nous débattons cette après midi me tient particulièrement à cœur. Je veux d’emblée dire ma satisfaction quant à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire : désormais, le code civil disposera que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

en effet, a le droit de jouir paisiblement de sa propriété, de son logement, de son fonds et d’obtenir réparation du préjudice qu’il subit. L’introduction de ce principe général dans le code civil consacre la jurisprudence de la Cour de cassation. Cela renforce la sécurité juridique du droit français et assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Le texte institue par ailleurs une exception tirée de la théorie dite de la « pré occupation », afin de trouver un meilleur équilibre entre les différents intérêts en présence. est posé le principe selon lequel celui qui s’installe à proximité d’un lieu particulièrement bruyant ou odorant ne peut se plaindre d’un trouble anormal du voisinage lorsque la nuisance existait déjà au moment de son installation. Le texte adopté par le Sénat en première lecture restreignait le périmètre de cette exception aux seules activités économiques. Je me félicite

Je salue également le travail de la CMP sur la notion d’installation du voisin lésé, qui figurait dans la proposition de loi initiale.

fait le Sénat en première lecture, de privilégier la référence à un acte juridique plutôt qu’à une notion de fait, sujette à interprétation. Je ne peux par ailleurs que me réjouir de la suppression bienvenue des deux alinéas relatifs aux troubles sonores des enfants, d’une part, et à la codification de la jurisprudence du Tribunal des conflits, Comme je l’avais dit devant vous en séance publique, les mots ont un sens. Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux les installations similaires ne sont pas, sauf cas extrême, des troubles anormaux de voisinage. Enfin, le Sénat a souhaité étendre le périmètre d’exonération des activités agricoles par l’ajout de dispositions spécifiques dans le code rural et de la pêche maritime. Il est en effet ubuesque que certains, dérangés par le bruit des tracteurs

la portée de cette exemption, le texte de la CMP vise l’hypothèse d’une modification non substantielle de la nature ou de l’intensité des conditions d’exercice de l’activité. Cette rédaction est plus prudente

le texte qui vous est soumis aujourd’hui est un texte d’équilibre et de concorde, comme l’a souligné la rapporteure. Il définit les contours de ce fameux « vivre ensemble », respectueux de chacun, que j’ai déjà évoqué devant vous. Cette avancée est permise par une rédaction issue d’un travail de compromis réalisé en parfaite intelligence par vos deux assemblées. Cette proposition de loi contribuera, j’en forme le vœu, dans le droit fil de la politique de l’amiable, à une résolution plus rapide des conflits et à la pacification des relations de voisinage sur l’ensemble du territoire – nous en avons grandement besoin

la proposition de loi, dans sa rédaction d’origine, découlait d’une réflexion de longue date autour de la codification du régime de la responsabilité sans faute du fait de troubles anormaux de voisinage. Cette notion juridique, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, repose sur l’appréciation du juge du fond, qui seul détermine la nature du trouble.

Ai je besoin de rappeler que les personnes les plus précaires sont souvent celles qui subissent les plus grands dommages liés à des troubles du voisinage, alors qu’elles n’ont pas de solution de relogement ? Les effets sur la santé de la fréquentation routière sont connus et entraînent des problèmes liés aux pollutions sonores et de l’air. La surfréquentation d’une route départementale liée à la création

Notre groupe, conscient des troubles liés à l’agriculture intensive, à l’industrialisation productiviste et au « quoi qu’il en coûte » économique, ne peut soutenir un tel texte. L’on peut et l’on doit prévoir un contrôle du juge sur les préjudices que subissent nos concitoyens du fait d’activités dans leur voisinage.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, si les conflits de voisinages ne sont pas nouveaux,

Je voudrais les remercier de jouer ce rôle de médiateur ou de conciliateur, qu’ils endossent parfois à leurs propres dépens. Il arrive en effet, malheureusement, que des maires soient agressés, parfois gravement, par des administrés, alors qu’ils tentent de régler des conflits de voisinage. Ils constituent le premier rempart contre ces phénomènes, et c’est bien souvent grâce à eux que de nombreux conflits de voisinage ne se judiciarisent pas. Nous ne pouvons les laisser seuls face aux maux de notre société. L’augmentation de ces conflits est symptomatique d’une dégradation du climat social et d’un affaiblissement du lien social dans notre pays. Dès lors, nous ne pouvons que saluer la volonté d’intégrer dans le code civil la notion de trouble anormal du voisinage. La codification proposée est une manière de garantir une application homogène de la jurisprudence sur tout le territoire. Il s’agit ici de légiférer sur l’obligation de réparer un dommage causé à son voisin. En la matière, nous devons prendre des précautions. Notre rôle est d’abord de trouver le juste équilibre entre la protection des personnes face à des voisins quérulents et la garantie du droit au recours pour les nombreuses victimes de nuisances anormales.

Il nous faut donc aussi agir pour que chacun ait droit à un environnement décent. Si nos usines et nos exploitations agricoles sont essentielles pour l’activité économique, il n’en reste pas moins que les personnes vivant à proximité des sites les plus polluants voient leur santé se dégrader,

populaire avoisinant. Si la maison mère américaine a été plusieurs fois condamnée pour pollution aux États Unis, cela n’a pas été le cas en France. Ne créons pas un droit à polluer, à faire du bruit et à détériorer la santé des plus précaires, au prétexte que cela faciliterait la réalisation de profits financiers. Il est de notre devoir de protéger l’intérêt général et de garantir un droit au recours à toutes les personnes victimes d’un trouble anormal de voisinage. Il ne saurait y avoir de sacrifiés de la pollution dans notre pays

nous devons aussi œuvrer pour l’intérêt général en retissant du lien social. Toutefois, nous voterons pour cette proposition de loi. La parole

Cette proposition de loi relative au régime de la responsabilité civile pour les dommages causés par les troubles de voisinage répond à des problématiques bien connues dans nos territoires. d’un côté, des entreprises, des associations culturelles ou sociales, qui font vivre nos territoires ; de l’autre, des habitants, qui cherchent à préserver leur cadre de vie. J’avais déjà évoqué, à cette tribune, le phénomène d’expansion des zones d’habitat, qui conduit au rapprochement géographique des zones d’activité économique et des habitations. Ce rapprochement entraîne inévitablement des frictions entre deux catégories d’occupants et une augmentation de la pression contentieuse sur les acteurs économiques. économiques. Des artisans ou des industriels sont obligés de renoncer à des projets, pourtant vertueux pour l’économie française. Ils sont même parfois contraints de partir.

extracontractuelle pour les préjudices du fait de troubles du voisinage. Je ne reviendrai pas sur l’importance des règles qui nous permettent de faire société et de bien vivre ensemble. Les débats que nous avions tenus dans cet hémicycle ont éclairé le texte que nous nous apprêtons à adopter. De la navette parlementaire sort un texte d’équilibre, qui répond à un double objectif : d’une part, un objectif de justice, qui passe par une conciliation entre les intérêts en présence, la liberté d’entreprendre et celle de jouir de ses biens d’autre part, un objectif de lisibilité du droit et, partant, de sécurité juridique, que ce soit pour les habitants ou pour les acteurs à l’origine des nuisances. C’est une avancée vers une meilleure prévisibilité de l’application du droit.

Comme l’a souligné Mme la rapporteure, cette rédaction permettra d’inclure notamment les activités associatives et culturelles, qui ne sont pas moins essentielles à la vie de nos collectivités. Je voudrais également saluer la solution équilibrée trouvée en CMP sur les troubles provenant des activités agricoles. Ce régime dérogatoire vient protéger les agriculteurs à deux titres, en sus de ce que prévoit le régime commun. D’abord, il prévoit une appréciation par le juge du caractère substantiel d’une modification de nature ou d’intensité de l’activité. Ensuite, et c’est le point principal, il protège les exploitants dans les cas où les nuisances seraient liées à une modification de l’activité ne visant qu’à se conformer aux lois et règlements. C’est une exigence : le poids de l’intérêt général exprimé dans les normes ne peut peser seulement sur quelques uns, surtout quand les conséquences préjudicielles peuvent être très lourdes. Si je m’inscris totalement dans la volonté de protéger nos agriculteurs, qui représentent une part importante de l’économie de nos campagnes, je voudrais tout de même réitérer mes regrets quant à la restriction de la dérogation au seul secteur agricole.

La ruralité ne désigne pas seulement un espace de repos, de loisir, de détente. C’est également un espace de production, de consommation et de développement. Nos concitoyens attendent de nous des perspectives et des garanties pour que ces territoires puissent continuer à produire et à se développer. Les habitants des villes, qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de s’établir durablement ou épisodiquement, lors des fins de semaine, dans ces territoires ruraux, aspirent de leur côté au calme et à la tranquillité. Ces attentes sont compréhensibles. Elles ne doivent toutefois pas porter préjudice aux projets et aux activités menés dans ces mêmes territoires. Le dialogue peut certes résoudre des incompréhensions et des crispations. Les agriculteurs et les industriels ont d’ailleurs bien souvent entrepris des efforts réels pour améliorer leurs relations avec leurs voisins. Néanmoins, les contentieux liés aux troubles de voisinage ont connu un essor préoccupant.

est aussi de nature à encourager les exploitants et les repreneurs, la transmission des exploitations étant un enjeu majeur dans la grande majorité des territoires.

groupe tient à réaffirmer que le maintien des sources de vitalité et de dynamisme dans nos territoires ruraux est non pas une option, mais une orientation ardente, légitime et bénéfique. Ce développement doit naturellement se concilier avec la vie de l’ensemble des habitants. La protection du voisinage, si elle constitue une exigence partagée, ne peut éclipser ou reléguer, sous n’importe quel prétexte, la liberté d’entreprendre, qu’elle soit agricole, industrielle ou associative.

nous voilà au terme de l’examen de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Derrière ces mots se cachent les troubles de voisinage dans une société contemporaine, qui prône le respect de l’autre et le vivre ensemble, mais qui bute au quotidien sur le délicat accommodement des hommes entre eux, sur la cohabitation parfois douloureuse de l’homme et de son environnement ou encore sur la difficile conciliation de l’activité humaine avec les activités économiques, agricoles, culturelles. Cette proposition de loi se donne donc pour objectif ambitieux de contribuer à l’apaisement de cette cohabitation. Malgré les efforts déployés, tant ici, au Sénat, qu’à l’Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire, force est de constater que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain reste encore et toujours circonspect quant à l’utilité de ce texte. l’avons dit : voilà près de quarante ans, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Il s’agit là d’un régime de responsabilité objective, objective, qui ne dépend pas de la démonstration d’un comportement fautif, mais qui requiert la démonstration d’un trouble permanent et continu, excédant la gêne normalement attendue dans le cadre des relations de voisinage. Celui ci peut être sonore, olfactif, esthétique, visuel, diurne, nocturne et s’exprimer en ville comme à la campagne. Il faut bien reconnaître qu’en quarante ans ce type de trouble n’a pas disparu. Pis, il s’en invente régulièrement de nouveaux : les poules, les tracteurs, la musique et même les enfants… Ce sont donc ces situations anciennes et nouvelles que la proposition de loi cherche à couvrir en ajoutant un nouveau chapitre au code civil intitulé : Les troubles anormaux du voisinage. et la spécificité des activités agricoles au travers d’un nouvel article du code rural et de la pêche maritime. Avec une telle articulation, les deux chambres pensent enfin avoir trouvé le bon schéma de cohabitation entre l’homme aspirant à sa quiétude et le développement d’activités utiles à notre société.

évidemment, les habitants aspirant à une vie à la campagne doivent entendre qu’il s’agit d’une vie de tous les jours et non pas de vacances. Et comme toute vie de tous les jours, celle ci peut être bruyante, odorante, parfois dérangeante. De même, les habitants préférant la vie en ville, parce qu’elle offre une foultitude de services et d’équipements, doivent entendre que ces aménités vont avec quelques effets secondaires comme les éclats de voix et de rire entendus depuis les trottoirs, les terrasses et les cours de récréation, ou encore le bruit des ballons qui rebondissent. Les élus que nous sommes savent que les Français, même s’ils restent très attachés à la défense des libertés collectives, sont aussi de plus en plus exigeants quant à leur liberté individuelle, à leur bien être ou à leur confort personnel. Cependant, aussi louable soit l’intention des auteurs de cette proposition de loi, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain n’est pas convaincu qu’elle arrivera véritablement à transformer certains voisinages disputés en paradis sur terre. Même si nous ne nions pas les efforts entrepris par les deux rapporteures pour surmonter leurs différences d’appréciation et pour chercher le nécessaire équilibre entre la liberté d’entreprendre et la protection de la jouissance d’un bien, entre la liberté d’installation et le droit au recours ou à réparation, je ne vous cache pas que nous ne sommes pas pleinement satisfaits du résultat de cette CMP conclusive. En effet, si la réécriture législative enrichit le code civil, il n’en reste pas moins qu’elle affaiblit le code de la construction et de l’habitation, et ce même si elle en garde l’esprit en englobant finalement toutes les activités,

décisions sur mesure que nos juges continueront de rendre plutôt que dans la capacité du code civil ou du code rural à dissuader froidement les requérants potentiels. Aussi, le doute subsistant, le groupe socialiste s’abstiendra sur ce texte. s’abstiendra sur ce texte. Pour améliorer notre vivre ensemble, la réponse la plus efficace du Gouvernement face à l’inquiétude du monde agricole et aux enjeux majeurs du logement et de la transition écologique serait plutôt de sécuriser les revenus et les investissements nécessaires. La

aux enjeux actuels dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Les troubles du voisinage constituent un problème récurrent. Nous sommes arrivés à un texte équilibré entre liberté d’entreprendre et protection de la jouissance d’un bien. Je souhaite saluer le travail de la rapporteure – chère Françoise Gatel –, qui a œuvré en ce sens. La rédaction finale répond à cette double exigence en reprenant les trois critères déjà établis, à savoir l’existence d’un dommage, l’anormalité du trouble et la relation de voisinage entre le défendeur et le demandeur. Bien que le droit en vigueur permette assez largement de répondre aux contentieux, la création d’un régime dérogatoire se justifie au regard de la nécessité de protéger nos territoires ruraux nos territoires ruraux et urbains face aux troubles anormaux de voisinage. Cette codification était attendue par de nombreux acteurs, en particulier les exploitants agricoles, essentiels au dynamisme économique et social de nos campagnes. Elle pourrait être jugée superfétatoire, mais c’est un signal opportun qui a son importance. Dans la rédaction finale, le terme générique « activités » permet de viser l’ensemble de ces dernières, qu’elles soient économiques, sociales, culturelles

l’objectif était de parvenir au meilleur équilibre possible entre, d’une part, la liberté d’entreprendre des agriculteurs et, d’autre part, le droit au recours et à la réparation d’un préjudice pour les voisins. La dérogation entérinée en commission mixte paritaire semble avoir atteint cet objectif.

Concernant le critère de la poursuite de l’activité, dès lors qu’une exploitation agricole modifierait les conditions d’exercice de son activité pour se mettre en conformité aux lois et règlements, le trouble anormal qui en résulterait ne pourrait engager la responsabilité de l’exploitant.

C’est le cas aujourd’hui avec cette proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Son article unique insère dans le code civil à la fois une création d’origine jurisprudentielle, à savoir la responsabilité sans faute en cas de trouble anormal de voisinage, et son exception, la théorie de la pré occupation. L’objectif est clair : limiter le nombre de contentieux de voisinage déclenchés par les personnes qui s’installent en milieu rural sans en accepter les particularités.

je me félicite de ce que la commission mixte paritaire ait été conclusive. L’esprit consensuel qui y a régné est la preuve de la ferme volonté de la représentation nationale de consacrer une jurisprudence bien établie,

À cet égard, je suis particulièrement heureux de souligner que les travaux du Sénat ont contribué à améliorer ce texte. Je veux parler de l’insertion dans le code rural d’une exonération particulière pour les activités agricoles. la responsabilité sans faute d’un exploitant agricole ne pourra pas être engagée si ses activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou si

Il faut protéger nos agriculteurs contre les actions abusives et aider les maires à désamorcer les conflits de voisinage au sein de leurs communes : la proposition de loi les aidera Quels sont ces avantages ? Elle permettra de contribuer à la pacification des relations de voisinage, à la ville comme à la campagne. Elle participera aussi au désengorgement des tribunaux

est question non pas de révolutionner le code civil, mais de le rendre plus lisible pour nos concitoyens. À l’issue de la CMP, il me semble que ce texte a atteint ces objectifs. Tout d’abord, il s’agit d’introduire dans le code civil le principe jurisprudentiel de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage afin d’en garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire national. Le texte prévoit également une exception tirée de la théorie de la pré occupation. Ainsi, une activité licite, antérieure à l’installation d’un nouveau voisin et continue ne saurait être contestée par ce dernier. Cette disposition répond aux préoccupations du monde rural de limiter les litiges avec les néoruraux. Je tiens à saluer les apports du Sénat et l’engagement sans faille de la rapporteure – chère Françoise Gatel. proposition de loi par la chambre haute a permis d’expliciter et de renforcer la protection des activités agricoles. À cet égard, vous avez obtenu une dérogation circonstanciée dans la cause exonératoire en faveur des activités agricoles. En commission mixte paritaire toujours, le Sénat a également permis de mieux préciser les critères d’installation. Un débat tout à fait légitime avait eu lieu dans cet hémicycle pour que les crèches et les écoles ne soient pas menacées de contentieux pour trouble anormal de voisinage. Les enfants pourront continuer de crier, puisque ce texte étend dans sa rédaction actuelle la dérogation à l’ensemble des activités, de quelque nature qu’elles soient. Par ailleurs, le caractère substantiel de modification d’activité restera opportunément soumis à l’appréciation souveraine du juge. Soyez rassurés, mes chers collègues, le recours au juge reste protégé par la Constitution. Les comportements que vous décriviez me semblent relever davantage du code de l’environnement, voire du code pénal. enfin à saluer la prise en compte des préoccupations légitimes exprimées dans les deux hémicycles. La commission mixte paritaire a permis de trouver un juste équilibre entre intérêt général, liberté individuelle et liberté d’entreprendre. offre une meilleure lisibilité aux justiciables, et ainsi une plus grande sérénité dans les rapports de bon voisinage, dont on sait à quel point ils sont primordiaux. En adoptant ce texte, nous ajouterons donc une modeste pierre à l’édifice d’un meilleur vivre ensemble. Le groupe Union Centriste votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Conformément Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Mes chers

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République du Kazakhstan Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge

j’ai l’honneur de présenter aujourd’hui le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre la République française et le royaume du Cambodge, signée à Paris le 26 octobre 2015 par les ministres de la justice des deux pays. La France et le Cambodge entretiennent une relation dynamique, qui a vocation à se renforcer encore davantage et à se diversifier. Cette relation est fondée sur des coopérations d’excellence, par exemple dans le domaine de la santé ou du patrimoine. La préservation du site d’Angkor illustre la richesse de ce travail commun. Les relations bilatérales avec le Cambodge se sont encore renforcées sous l’impulsion du Président de la République. Le Cambodge adhère aux ambitions de l’accord de Paris ; il pourra compter sur la France comme partenaire sur les enjeux globaux. globaux. Nos deux pays partagent une communauté de valeurs, notamment un attachement à la Charte des Nations unies. Cet attachement s’est matérialisé par la prise de position du Cambodge à l’Assemblée générale des Nations unies

La France, coprésidente de la conférence qui a conduit à la signature des accords de paix à Paris, le 23 octobre 1991, y veille avec une attention particulière. Ces accords appellent le royaume du Cambodge à mettre en œuvre les mesures qui permettront d’assurer une réelle démocratie, pluraliste et respectueuse des libertés fondamentales. Pour ces raisons, et au regard de la dynamique de notre relation et du rôle historique de la France, nous avons avec le Cambodge un dialogue franc et constructif sur la question de la démocratie et des droits de l’homme. Nous n’éludons aucun sujet. Nous n’avons ainsi pas hésité à déplorer les mesures restrictives à l’encontre de médias indépendants et de membres de l’opposition dans les mois qui ont précédé les élections législatives de 2023. Le Cambodge sait que le renforcement de notre partenariat suppose de veiller au respect des droits de l’homme. La convention d’extradition soumise à votre approbation est une illustration de la dimension opérationnelle de cette coopération. Ce texte vient compléter le tissu conventionnel avec ce pays dans le domaine judiciaire, la France et le Cambodge étant d’ores et déjà partie à plusieurs conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations unies la convention unique sur les stupéfiants, adoptée en 1961 ; la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1984 la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée en 1988 ; la convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en 2000 ; la convention contre la corruption, adoptée en 2003. Cependant, aucune convention bilatérale ne lie nos deux pays en matière de coopération judiciaire. La coopération en matière d’extradition repose actuellement sur le principe de réciprocité dans le cadre de la courtoisie internationale. Depuis le 1 janvier 2009, quatre demandes d’extradition ont été échangées entre la France et le Cambodge : trois ont été émises par les autorités françaises, une par les autorités cambodgiennes. Les demandes d’extradition émises par la France ont concerné des faits de viol sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles aggravées, trafic de stupéfiants, abus de confiance, escroquerie, faux et blanchiment. Elles avaient pour fondement tant des poursuites que l’exécution d’une peine. Toutes ces demandes ont donné lieu à la remise de la personne recherchée. recherchée. L’unique demande d’extradition passive a quant à elle donné lieu à un avis défavorable de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris en raison du caractère incomplet des réponses apportées par le gouvernement cambodgien. la convention qui est aujourd’hui soumise à votre approbation a pour double objectif de faciliter et d’encadrer les demandes d’extradition entre nos deux États. Elle énonce un engagement d’extradition fondée sur une infraction pénale ou une condamnation pénale comportant une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l’autre partie à la suite d’une infraction pénale. Cependant, la convention prévoit plusieurs motifs de refus obligatoires ou facultatifs. Ainsi, l’extradition ne sera pas accordée lorsque la partie requise considère que la personne recherchée est réclamée pour une infraction politique ou encore lorsqu’elle a des raisons sérieuses de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations d’origine ethnique, de sexe, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. En outre, conformément au principe de respect des droits de la défense, une demande d’extradition sera rejetée si la personne réclamée doit être jugée dans la partie requérante par un tribunal d’exception n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure doit exécuter une peine infligée par un tel tribunal. L’extradition sera également refusée si les faits qui la motivent sont passibles de la peine de mort. cependant à rappeler que la peine de mort a été abolie au Cambodge en 1989. Je sais que plusieurs sénateurs ont émis en commission des réserves sur cette convention, fondées sur une inquiétude en matière de respect des droits de l’homme. messieurs les sénateurs, cette question a bien été intégrée et les dispositions de la convention sont protectrices des droits et libertés fondamentales. Pour conclure, il convient de relever que le royaume du Cambodge a ratifié cette convention le 14 octobre 2020. Telles sont, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle la convention d’extradition signée en 2015 avec le royaume du Cambodge, qui fait l’objet du projet de loi aujourd’hui soumis à votre approbation. La parole

Le royaume du Cambodge a, pour sa part, achevé la ratification de cette convention depuis le 14 octobre 2020. Précisons le d’emblée, il est manifeste que l’enjeu de ce texte ne se limite pas à sa portée opérationnelle,

Ces échanges extraditionnels, jusqu’à présent réalisés sur le fondement d’un principe informel de réciprocité, se trouvent tributaires du bon vouloir des parties ; leur sécurisation juridique pâtit de cette absence de cadre formel. Cependant, compte tenu de leur caractère sporadique, la signature d’une convention bilatérale ne s’imposait pas vraiment d’un point de vue strictement opérationnel. C’est pourquoi, au cours de sa réunion du 6 mars dernier, c’est sur le double contexte dans lequel s’inscrit ce texte que la commission des affaires étrangères a essentiellement débattu

la Constitution comme la loi pénale cambodgiennes garantissent le respect des droits de l’homme, la liberté d’expression, l’indépendance des juges, la séparation des pouvoirs, les droits de la défense, la présomption d’innocence et encadrent strictement la garde à vue et la détention provisoire. il est clair que la mise en pratique de cette panoplie de garanties, qui n’a rien à envier aux démocraties les plus abouties, n’est pas à la hauteur des principes affichés.

et dissolution de son parti ; condamnation par contumace de Sam Rainsy et de soixante dix autres opposants à des peines allant de vingt ans de prison à la perpétuité ; diverses mesures entravant le droit de vote et la liberté de la presse… Les syndicalistes, les défenseurs des droits fonciers, les militants écologistes font également l’objet d’intimidations et d’arrestations, que les ONG dénoncent régulièrement. Cette situation interne a valu au royaume du Cambodge de se voir retirer par l’Union européenne, dès 2020, une partie des préférences commerciales qui lui avaient été accordées au titre du régime « Tout sauf les armes » (TSA), dont il bénéficiait depuis 2001.

la commission a jugé rassurantes les garanties apportées aux justiciables par le texte. Sa rédaction, qui reprend le texte proposé par la France, est conforme en tous points aux standards juridiques nationaux et internationaux. Les motifs de refus qu’elle prévoit – les infractions politiques, les demandes paraissant motivées par l’origine ethnique, le sexe, la nationalité ou la religion de la personne réclamée, ainsi que le fait de posséder la nationalité de la partie requise – entraînent le rejet immédiat du dossier et interdisent toute demande d’extradition abusive ou formulée à l’encontre d’un opposant au régime. la commission a observé qu’alors même que la peine capitale a été abolie au royaume du Cambodge en 1989 et que sa prohibition est inscrite dans sa constitution depuis 1993, la convention prévoit fort prudemment une clause de substitution de cette peine, afin de parer à toute tentation de retour en arrière. Enfin, une clause dite humanitaire permet de rejeter une extradition susceptible de mettre en danger la personne réclamée en raison de son âge ou de son état de santé, ce qui nous est également apparu tout à fait pertinent. Cet arsenal de précautions constitue autant de garde fous qui encadrent la mise en œuvre de la future convention. La commission des affaires étrangères a estimé que, dans ces conditions, rien ne s’opposait à opérer, en cas de besoin, des échanges extraditionnels avec le royaume du Cambodge,

informel de réciprocité, n’en seront que mieux cadrées et sécurisées, tant sur le fond que sur la forme. Le second élément de contexte qui a nourri nos échanges en commission lors de l’examen de cette convention est la relation bilatérale franco cambodgienne.

avec la visite officielle de Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, au mois de novembre 2023, et celle du nouveau Premier ministre Hun Manet, le 18 janvier dernier. À cette occasion, les dirigeants cambodgiens ont réaffirmé leur volonté d’approfondir cette relation et se sont montrés demandeurs d’un partenariat renforcé avec la France. Ces contacts récents s’inscrivent dans la continuité d’une coopération de longue date, héritée à la fois d’une histoire commune et du rôle central joué par la France dans le développement du pays et dans la mise en place de ses institutions, depuis les accords de Paris de 1991. La présence très active de la communauté cambodgienne en France et la place importante de la francophonie au sein du royaume contribuent à nourrir ces liens. Il y a donc une logique historique au renforcement de notre partenariat, à laquelle notre commission a été sensible.

De plus, cette relation privilégiée peut constituer un cadre efficient pour accompagner des évolutions positives dans le domaine des droits de l’homme, notamment au regard de la lutte contre l’impunité, de la question de l’égalité des droits des personnes LGBT+, du droit de l’environnement, ou pour œuvrer en faveur de la grâce d’opposants au régime. Tel est le sens que je souhaite donner à l’adoption de ce projet de loi, qui a été approuvé par la commission des affaires étrangères dans sa majorité : un regard sans naïveté ni complaisance sur la situation intérieure du royaume, mais aussi le choix d’approfondir notre relation bilatérale avec un pays qui se trouve à la croisée des chemins, entre une influence chinoise particulièrement présente et une volonté de cultiver ses liens avec la France en renforçant et en diversifiant un partenariat ancré dans notre histoire commune.

convention qui attend sa ratification depuis 2015. En effet, depuis sa signature par Mme Taubira, alors garde des sceaux, ce texte a été déposé trois fois à l’Assemblée nationale ou au Sénat ; à chaque fois, il a fini par être retiré. Ces rétropédalages successifs sont liés à la détérioration très préoccupante de la situation des droits de l’homme dans le royaume du Cambodge.

Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Cambodge a par ailleurs fait état, dans son rapport en date du 20 juillet 2023, d’arrestations et de poursuites injustifiées à l’encontre de défenseurs des droits humains, de journalistes ainsi que de dissidents politiques. Notons par ailleurs que le parti du sauvetage national du Cambodge, principale formation d’opposition, reste interdit et que les actions engagées contre ses membres et les militants du parti de la bougie, qui lui a succédé, se poursuivent encore aujourd’hui. D’ailleurs, cette situation a conduit l’Union européenne à retirer dès 2020 une partie des préférences commerciales accordées au Cambodge au titre du régime « Tout sauf les armes », dont il bénéficiait depuis 2001. En outre, l’augmentation considérable de la population carcérale et les conditions de vie dans les prisons du pays sont pointées par ces différents rapports.

Les observations finales concernant le troisième rapport périodique du Cambodge, publié le 18 mai 2022, sont plus préoccupantes encore. si le Comité des droits de l’homme se félicite que les droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques soient traduits dans la législation, il s’est tout de même déclaré profondément préoccupé par les graves allégations de tortures et de mauvais traitements infligés en garde à vue et dans d’autres lieux de détention. Dès lors, après lecture de ces différents rapports, soutenir la ratification de cette convention, c’est, une fois de plus, signer un « deux poids, deux mesures » en matière de défense et de respect des droits humains. Ce double standard ulcère légitimement nos concitoyens et décrédibilise la voix de la France sur la scène internationale. C’est pourquoi nous pensons nécessaire de voter contre ce texte tant que nous n’aurons pas de solides garanties montrant la fin de telles exactions contre les droits humains.

Cependant, pour une meilleure sécurisation juridique de l’extradition, cet arsenal multilatéral mérite d’être complété par une coopération bilatérale directe. Aussi

Malgré la faiblesse du nombre de cas potentiellement concernés, cette convention d’extradition entre nos deux pays permettra de renforcer la lutte commune contre la criminalité. Enfin, cette convention répond à une exigence plus globale d’adaptabilité de la coopération judiciaire, au regard d’enjeux autour de litiges transnationaux, majoritairement d’ordre intrafamilial, ou de la question de l’exploitation sexuelle. évidemment, nos débats sur ladite convention ne doivent pas occulter la situation très fragile des droits de l’homme dans ce pays, ainsi que la dérive autoritaire du régime. À ce titre, le haut commissaire aux droits de l’homme des Nations unies a qualifié la situation démocratique du pays de « très préoccupante Lors des élections législatives du mois de juillet dernier, les partis d’opposition, les syndicats et les médias ont été ciblés par des procédures judiciaires, des intimidations et, parfois, des menaces physiques… Ne pas retenir la procédure d’examen simplifié pour ce texte sert la vigilance, dont notre assemblée doit faire preuve. C’est également l’occasion de rappeler la nécessité pour nos entreprises françaises de ne pas contribuer au désordre environnemental qu’engendre la stratégie dite du pentagone, mise en place par le Premier ministre cambodgien. De jeunes militants écologistes sont jetés en prison parce qu’ils défendent les forêts cambodgiennes, menacées par des projets économiques d’envergure. Par ailleurs, le Vietnam s’inquiète du grand risque de désastre écologique qu’entraînerait le détournement des eaux du Mékong projeté par son voisin. Au delà de ces exigences, on ne peut nier la nécessité de conserver le dialogue avec le pouvoir en place, dans un contexte et une région du monde en proie aux velléités impérialistes de l’axe sino russe. Dès lors, nous considérons que cette convention s’inscrit dans une dynamique de rapprochement de nos deux pays, au nom de la stabilité régionale. Les récents échanges diplomatiques entre le président Macron et le roi Norodom Sihamoni, puis le Premier ministre cambodgien, illustrent les efforts déployés pour renforcer nos relations bilatérales.

RDSE se réjouit de ce rapprochement, qui s’inscrit en effet dans la stratégie indo pacifique de la France, mais sans perdre de vue les efforts que Phnom Penh doit fournir en matière démocratique pour arriver à un niveau de responsabilité satisfaisant. Espérant que ce projet de loi y contribuera, même modestement, le groupe RDSE l’approuvera. La parole

Depuis lors, le projet de loi d’approbation de ladite convention a connu un parcours difficile, symptôme des remous diplomatiques qui ont animé les relations entre la France et le Cambodge. Celles ci se stabilisent, comme en témoigne la rencontre entre le Président de la République et le Premier ministre du royaume du Cambodge, le 18 janvier 2024. Voilà donc l’occasion pour notre Parlement de débattre enfin sur ce texte, qui a été déposé, puis systématiquement retiré à plusieurs reprises entre 2016 et 2022. Aboutissement des négociations bilatérales entre la France et le Cambodge, cette convention entend permettre le renforcement de la coopération entre les deux pays. Son approbation serait également un pas de plus vers la concrétisation du projet de convention d’entraide en matière pénale, second aspect des négociations entre la France et le Cambodge.

Alors ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, M. Olivier Becht affirmait au mois de janvier 2023 que la relation économique entre la France et le Cambodge était déjà forte, mais qu’elle pouvait se renforcer davantage. Ce souhait est toujours d’actualité, les chefs d’État français et cambodgien ayant depuis réitéré leur souhait de voir les investissements bilatéraux fleurir et les partenariats économiques se renforcer. J’ai souhaité rappeler le rôle géopolitique et économique qu’occupe le Cambodge pour souligner l’importance d’une bonne entente et d’une coopération solide entre ce pays et le nôtre. N’oublions pas que nous partageons une histoire et des valeurs communes. La France souhaite que le Cambodge soit représenté à haut niveau au XIX sommet de la francophonie, au mois d’octobre prochain. Le Cambodge fait par ailleurs preuve d’exemplarité en matière de promotion de la francophonie : le pays a officialisé son souhait d’accueillir la XX édition de ce sommet en 2026. En matière environnementale, nous partageons et nous soutenons l’ambition cambodgienne d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Par ailleurs, les liens culturels et historiques qui lient nos deux pays sont de toute évidence très forts et inaltérables. Notre histoire commune s’écrit en français et en cambodgien. Poursuivre l’écriture de cette histoire à deux plumes nécessite de voter le présent projet de loi et d’approuver définitivement la convention d’extradition qui erre dans les limbes législatifs depuis trop longtemps. Au delà du contexte politique et géopolitique dont nous avons déjà discuté, concentrons nous sur le texte en lui même. La convention comprend des dispositions importantes et poursuit un but vertueux, à savoir le renforcement des capacités communes de la France et du Cambodge dans la recherche et l’appréhension de malfaiteurs en fuite. Le Cambodge, où continue malheureusement de prospérer le trafic d’êtres humains, notamment des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle, peut être un pays refuge pour des Français auteurs d’infractions à caractère sexuel. Que dire, à part que cette convention est un pas dans la bonne direction pour assurer l’extradition de ces malfaiteurs, la bonne tenue de leurs procès et, le cas échéant, la bonne application de la peine qui en résultera ? Enfin, je tiens à préciser que je respecte mes collègues qui s’inquiètent des manquements cambodgiens en matière de droits de l’homme, de la liberté de l’information et du pluralisme politique. Ces manquements sont indéniables et les inquiétudes exprimées sont toutes légitimes. que l’histoire récente laisse entrevoir une évolution positive du Cambodge sur de nombreux sujets. Dans leur déclaration commune faisant suite à leur entretien du mois de janvier dernier, le Président de la République et le Premier ministre cambodgien ont tous deux reconnu la nécessité du pluralisme politique et la protection des droits fondamentaux, deux piliers de la démocratie. Ils ont tous deux exprimé leur souhait de coopérer en ce sens. Cette nette amélioration des relations entre la France et le Cambodge s’accompagne du témoignage de la bonne volonté du Cambodge dans le respect

les relations étroites et si singulières tissées au fil du temps, l’amitié réelle et la considération mutuelle que cultivent nos deux pays, mais aussi les mémoires collectives imprégnées de moments souvent insoutenables ont cette capacité à atténuer la distance géographique qui sépare Phnom Penh de Paris. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement naturel de ce long mouvement de rapprochement entre nos deux peuples. Deux peuples qui cultivent leur attachement à la langue française, une communauté francophone forte de 463 000 locuteurs Deux peuples qui ont fait le choix de conforter les coopérations économiques, culturelles, éducatives ou encore militaires et de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales depuis 2022. Deux peuples qui ont inscrit au plus haut de leur hiérarchie des normes les valeurs de démocratie et de liberté. En effet, en 1993, après des décennies de conflits et de régimes autoritaires, la promulgation de la Constitution cambodgienne a eu vocation à engager le pays sur le chemin de la démocratie. La loi fondamentale proclame ainsi la séparation des pouvoirs et un certain nombre de droits et de libertés, notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et le droit à un procès équitable : autant de valeurs dans lesquelles la France se reconnaît. Au delà de ces principes, au delà du texte, la situation est en réalité bien plus contrastée dans ce pays, où la vie politique est dominée par le parti du peuple cambodgien, dirigé depuis 2015 par l’ancien Premier ministre Hun Sen, dont le fils Hun Manet a récemment pris la tête du gouvernement. Au delà des proclamations, la liberté est trop souvent atrophiée par un régime qui a privé les dernières élections de toute opposition crédible. Au delà des intentions, l’arbitraire est désormais enraciné dans cet État, qui ordonne la fermeture de son dernier titre de presse indépendant, qui multiplie les intimidations et les arrestations et dans lequel la corruption s’enkyste. C’est précisément pour ces raisons que le débat que nous avons aujourd’hui me semble nécessaire. Je veux d’ailleurs saluer mes collègues parlementaires qui ont pris l’initiative de ce texte, le retour à la procédure normale. Ce débat constitue l’occasion pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain de dénoncer les atteintes préoccupantes aux droits humains, qui ternissent l’image du Cambodge depuis 2017 – ce qu’il fait à cet instant avec clarté. Ce débat nous permet également d’évoquer cette histoire commune et ces liens étroits avec le Cambodge, qui nous conduisent, en responsabilité et avec précaution, à favoriser un approfondissement des relations bilatérales avec ce pays. Sur ce point, monsieur le rapporteur, nous faisons le même constat que vous, celui d’une nouvelle dynamique à l’œuvre dans le cadre des relations bilatérales qu’entretiennent nos deux États. Cela s’est confirmé avec la visite de travail du Premier ministre Hun Sen en France à l’hiver 2022, puis avec celle du roi du Cambodge à l’automne dernier et, plus récemment encore, avec celle du nouveau Premier ministre, Hun Manet, reçu par le Président de la République en début d’année. Oui, la France doit aller plus loin dans sa relation avec le Cambodge. Mais le chemin de la coopération ne peut être emprunté sans poser des garanties claires et sans déterminer une direction commune, celle du confortement de nos démocraties. concerne les garanties, la convention soumise à notre examen peut être qualifiée de « robuste » au regard des précautions qu’elle comporte. Comme cela a déjà été souligné, le texte prévoit un certain nombre de garde fous. Je veux à ce titre souligner qu’il s’inspire largement des dispositions de la convention européenne d’extradition de 1957. Cette convention avec le Cambodge détaille par ailleurs les motifs de refus parmi lesquels les infractions de nature politique ou militaire. N’entrent pas non plus dans le champ de cet accord les demandes motivées par des considérations d’origine ethnique, de sexe, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques. parce que nous savons que la quasi totalité des opposants au régime qui sont réfugiés en France possèdent la double nationalité, la convention les préserve de toute demande d’extradition. Ce texte permet donc de renforcer les capacités communes de nos deux États dans la recherche et l’appréhension des malfaiteurs en fuite. Il confortera notre coopération en matière de lutte contre la criminalité tout en garantissant la préservation de libertés fondamentales face à l’arbitraire et aux abus de pouvoir. Concernant la direction que nous voulons prendre, je voudrais vous faire part d’une conviction : oui, le dialogue avec d’autres États peut contribuer à faire rayonner les valeurs universalistes que nous promouvons. Et c’est précisément à ce titre que nous demandons au Gouvernement de faire de cette convention un outil complémentaire au service du rapprochement entre la France et le Cambodge et de faire du resserrement de ces liens et du dialogue bilatéral un moyen de tendre vers une évolution positive de la situation des droits humains dans ce pays. Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement doit continuer d’inscrire à l’ordre du jour de ses échanges avec les autorités cambodgiennes la question du rétablissement et de la préservation des libertés publiques. La France doit La France doit également poursuivre son rapprochement avec le Cambodge afin de faire progresser nos valeurs communes. En votant pour l’approbation de cette convention d’extradition, nous faisons le pari de l’avenir, en responsabilité, avec la lucidité et la vigilance que celle ci exige. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain suivra donc l’avis de la commission, avec les réserves que je viens d’évoquer.

Au fil de ce riche passé commun, se sont développés entre nos deux nations des affinités profondes ainsi que de véritables liens d’amitié, de respect et de confiance mutuels. Ces liens amèneront notamment la France à assumer un rôle de premier plan dans les accords qui, en 1991, permirent au peuple cambodgien de tourner enfin la page la plus tragique de son histoire contemporaine, après deux décennies de folie khmère rouge et de guerre civile meurtrière. Aujourd’hui, les relations franco cambodgiennes demeurent étroites. Elles s’épanouissent dans une volonté partagée de faire vivre une francophonie dynamique et dans le souhait de développer des liens économiques structurés non seulement par les investissements de nos grands groupes, mais aussi par la présence sur place de nombreux entrepreneurs français. Nos relations se déploient également dans divers autres secteurs. Elles s’appuient sur une aide au développement conséquente, sur des échanges universitaires nourris – en particulier dans le domaine de la santé –, sur des contacts fructueux au niveau militaire et sur des coopérations dans l’éducation, le le changement climatique, la biodiversité ou encore la culture et le patrimoine, au travers notamment des actions menées pour la sauvegarde du fabuleux site d’Angkor. Récemment, nos deux pays se sont engagés dans la voie d’un renforcement de ce partenariat. Dans le contexte géopolitique actuel, chacun y trouve en effet un intérêt bien compris. La zone indo pacifique, qui concentre certaines des routes commerciales les plus empruntées au monde, représentera en 2040 plus de la moitié du PIB mondial et constituera, à ce titre, la principale réserve de la croissance globale des années à venir. La région attire donc autant les convoitises qu’elle cristallise les tensions, en particulier entre une Chine aux volontés de plus en plus hégémoniques et des États Unis de plus en plus soucieux de contrer Pékin partout où ils le peuvent. Pour la France, puissance riveraine de l’Indo Pacifique par ses outre mer, un réengagement solide dans la région est essentiel et le Cambodge peut représenter un point d’appui important. Quant à nos partenaires cambodgiens, ils perçoivent dans l’offre française, qu’ils savent coopérative et inclusive, un moyen de diversifier leurs partenariats et de desserrer un peu l’omniprésence économique de la Chine sans pour autant se retrouver pris en étau dans la rivalité sino américaine. La convention d’extradition que nous examinons s’inscrit donc comme un jalon sur le chemin de ce rapprochement stratégique voulu à la fois par Paris et par Phnom Penh. Négociée sur l’initiative de notre pays et signée en 2015, elle vient enrichir la relation dans un domaine où nous ne sommes liés par aucun accord bilatéral et où la coopération est menée sur une base, sans autre cadre que celui posé par les conventions multilatérales. Ce texte ne soulève pas en soi de problème particulier. En premier lieu, parce qu’il ne devrait concerner qu’un nombre limité de cas au vu du très faible volume de demandes d’extradition formulées par la France et le Cambodge au cours des quinze dernières années. Ensuite, parce qu’il s’agit d’un accord conforme aux standards internationaux en la matière, semblable aux multiples conventions de cette nature signées par la France avec d’autres pays. Ce texte dispose donc de toutes les garanties procédurales nécessaires à la prévention d’éventuels abus. À cet égard, je pense tout particulièrement aux dispositions encadrant les motifs de refus des extraditions. Ces dernières devront récusées si elles concernent des infractions militaires, mais aussi – et surtout – des infractions politiques. Si ces dispositions revêtent une importance aussi prégnante, c’est naturellement en raison de la situation au Cambodge.

Si le Cambodge a ratifié la plupart des conventions internationales sur les droits de l’homme, s’il a formellement mis sa législation en conformité avec ses engagements et s’il a – cela mérite d’être souligné – constitutionnalisé l’abolition de la peine de mort dès 1993, la réalité n’en est pas moins que les opposants politiques, les responsables syndicaux ou les journalistes font l’objet de nombreuses pressions, quand ils ne sont pas tout simplement incarcérés et leurs organisations interdites. La situation avait ainsi conduit l’Union européenne, avec le soutien de la France, à suspendre en 2020 le traitement préférentiel accordé à Phnom Penh dans le cadre du régime commercial « Tout sauf les armes ». La question du respect des droits de l’homme est donc une préoccupation tout à fait centrale. Toutefois, en la matière, la voie du dialogue – un dialogue certes exigeant – me semble toujours préférable à celle de l’ostracisme. C’est la méthode la plus efficace pour accompagner les évolutions positives que nous appelons tous de nos vœux. Or cette volonté de dialogue rencontrera une oreille d’autant plus attentive qu’elle sera exprimée dans le cadre d’une relation bilatérale solide et approfondie. En outre, l’arrivée au pouvoir, l’année dernière, de Hun Manet peut constituer une occasion à saisir. Bien évidemment, on ne peut ignorer que cette succession est avant tout de nature dynastique, puisque le nouveau Premier ministre n’est autre que le fils de son prédécesseur, resté trente huit ans au pouvoir. Il ne faut donc pas se bercer d’illusions et imaginer que le Cambodge pourrait du jour au lendemain s’engager sur la voie d’un changement complet de régime et adopter en la matière les pratiques qui sont les nôtres. Néanmoins, l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants déterminés à réformer et à développer leur pays et demandeurs, à cette fin, d’une relation renouvelée avec le nôtre, installe un contexte favorable pour que la voix de la France porte davantage, y compris sur la question fondamentale des droits civils et politiques. C’est donc en formant ce vœu pour les années à venir que le groupe Les Républicains, suivant en cela la recommandation de la commission des affaires étrangères, se prononcera en faveur de l’approbation de cet accord conclu avec le royaume ami

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ces dernières années, Phnom Penh s’est montrée désireuse de se rapprocher de Paris, tant pour accroître son développement que pour équilibrer quelque peu l’énorme influence du voisin chinois. Depuis janvier dernier, la France est devenue le quatrième partenaire stratégique du Cambodge aux côtés du Japon, de la Chine et de la Thaïlande. Nous avons ainsi la chance d’accompagner le développement cambodgien. Nos entreprises peuvent utilement contribuer à la construction et à la modernisation des infrastructures de ce pays. l’Association des nations de l’Asie du Sud Est (Asean), l’un des centres économiques majeurs du monde. Il est important que la France puisse y faire entendre sa voix. Au delà des opportunités économiques et commerciales que représentent cette relation, notre coopération concerne également le domaine de la défense. L’année 2023 a marqué la poursuite d’un rapprochement avec le Cambodge, dont nous ne pouvons que nous féliciter. Il intervient à la faveur d’une évolution politique dans le pays et s’inscrit dans la vision de l’Indo Pacifique développée par le Président de la République. Nous ne devons – ni ne pouvons – nous désintéresser de cette région du monde : les enjeux y sont trop importants et nous y avons des intérêts à défendre. Le texte que nous examinons vise à ratifier un accord de coopération judiciaire entre nos deux pays, comprenant notamment un dispositif d’extradition. La France a tout intérêt à ce renforcement des liens avec le Cambodge, mais cette coopération ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Nous ne pouvons transiger sur nos valeurs les plus essentielles. Nos deux pays sont liés par une longue histoire. Au cours de celle ci, ils se sont tantôt éloignés, tantôt rapprochés. La France a plusieurs fois protesté contre les atteintes aux droits de l’homme commises dans le royaume. La législation de ce pays a néanmoins évolué vers une meilleure protection des libertés individuelles, qu’il reste encore à traduire dans les faits. Ces progrès récents nous permettent cependant d’envisager plus sereinement l’avenir de notre coopération. Il nous semble donc que le processus de ratification doit être relancé, et ce d’autant plus que les accords et les échanges sont un moyen efficace de promouvoir nos principes. Nous ne pouvons pas attendre que le monde devienne conforme à nos idéaux – cela vaut ici comme ailleurs. Nous devons travailler dès aujourd’hui à le rendre meilleur. La coopération en matière judiciaire est un sujet particulièrement sensible. Tout d’abord, la lutte contre la criminalité est essentielle pour établir l’État de droit. Ensuite, nous souhaitons nous prémunir contre toute instrumentalisation des procédures. À cet égard, l’accord conclu encadre strictement cette coopération et prévoit une série de garanties permettant de prévenir d’éventuelles dérives. Nous devons encourager les évolutions qui sont à l’œuvre dans le Cambodge moderne. Le groupe des indépendants soutient par conséquent l’adoption de ce projet de loi tout en appelant le Gouvernement à la plus stricte vigilance sur la question des droits humains.

des liens indéfectibles unissent la France et le Cambodge. Ces liens, forgés au fil des siècles, sont le fruit d’une histoire commune, parfois complexe, mais toujours empreinte d’un profond respect mutuel. mutuel. Nous ne sommes pas appelés aujourd’hui à prendre position sur les liens d’amitié entre nos deux nations. Nous devons nous positionner sur un projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Cambodge. Nous devons le faire non seulement en tant que sénateurs, mais aussi en tant que défenseurs des droits humains et de la dignité humaine. Or l’amitié entre nos deux peuples nous oblige à tenir un discours de vérité. La convention d’extradition récemment signée entre la France et le Cambodge, bien qu’elle marque un progrès en matière de coopération judiciaire,

de violence, d’abus et même de mort en détention soulignent un manquement grave aux principes fondamentaux des droits humains. Ce n’est pas seulement une question de politique intérieure cambodgienne ; c’est une question qui doit interpeller notre conscience et qui doit rejaillir, par extension, sur notre coopération bilatérale avec le Cambodge en matière d’extradition. Comment pouvons nous assurer la protection des droits fondamentaux à des personnes extradées vers des prisons où la torture et les traitements inhumains sont rapportés comme étant des pratiques courantes dans le cadre de la lutte contre la drogue ? Il est crucial de rappeler que le Cambodge a aboli la peine de mort et inscrit la prohibition de cette peine dans sa Constitution. C’est un pas en avant pour les droits humains. Cependant, les actes de torture et les conditions déplorables de détention nous poussent à nous interroger sur l’effectivité de ces engagements constitutionnels. Face à cette situation, nous, élus du groupe écologiste, proposons que la France adopte une position ferme et claire en matière de coopération avec le Cambodge. En tant que Nation, nous portons la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits humains, non seulement à l’intérieur de nos frontières, mais également dans le cadre de nos relations internationales. Ce n’est qu’en adoptant une approche cohérente et engagée en matière de droits humains que nous pourrons contribuer à l’édification d’un monde plus juste et plus humain. Les liens historiques et d’amitié entre le peuple français et le peuple cambodgien sont un héritage précieux que nous devons continuer à cultiver et à développer. Ce sont justement ces liens d’amitié qui nous permettent de dire les choses avec franchise. nous voterons contre ce projet de loi. Nous espérons toutefois que nous saurons trouver ensemble, avec nos amis cambodgiens, la voie d’une coopération respectueuse du droit des peuples et des droits fondamentaux tout en gardant à l’esprit l’importance de notre rôle en tant que défenseurs de la dignité humaine dans nos rapports avec nos partenaires internationaux. La discussion

aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Cambodge. Mes chers

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je veux réaffirmer à cette tribune le caractère hautement stratégique d’EDF pour notre pays, en tant qu’opérateur historique.

France » –, cette proposition de loi a été grandement transformée au cours de nos discussions. Elle l’a tout d’abord été grâce à l’action du Gouvernement, qui a agi promptement pour protéger le groupe Électricité de France. L’offre publique d’achat simplifiée qu’il a lancée en 2022 a été un succès : le capital d’EDF est désormais détenu à 100 % par l’État.

L’accès aux TRVE des nombreux boulangers, restaurateurs ou fleuristes qui en étaient exclus jusqu’alors renforcera les tissus économiques et sociaux locaux et les protégera en cas de nouvelle crise énergétique.

Nous pensons qu’il constitue désormais un texte raisonnable, réaliste et utile, pour protéger tant le groupe EDF que les TPE

nationale. Si, à l’évidence, ce texte a considérablement évolué et si d’aucuns peuvent regretter le redimensionnement de son contenu, je pense néanmoins que nous pouvons être collectivement fiers du travail mené par l’ensemble des parlementaires.

de retrouver le contrôle de notre souveraineté énergétique et de protéger les Français contre la précarité énergétique qui les accable. Tous ces enjeux d’intérêt supérieur rendaient impératifs un dialogue et donc un compromis : c’est la méthode que nous avons tous scrupuleusement appliquée.

Sans avoir pour objectif de figer définitivement la structure capitalistique d’EDF, cette rédaction impose au Gouvernement de saisir le Parlement pour toute nouvelle évolution de la participation publique au capital de la société.

le réarmement du service public de l’électricité est devenu une urgence du temps présent et un impératif pour notre avenir. C’est la raison pour laquelle, au delà de cette proposition de loi, nous demandons de nouveau au Gouvernement de définir une stratégie claire

sans condition de puissance souscrite à l’ensemble des très petites entreprises et des collectivités dont le budget s’élève à moins de 2 millions d’euros et comptant moins de dix équivalents temps plein. Face à la volatilité des prix de l’énergie, il s’agit d’un bouclier vital pour nos millions d’artisans, de commerçants, de restaurateurs et d’agriculteurs. je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous auront permis de nous rassembler autour de choix stratégiques pour assurer la souveraineté et l’indépendance de notre pays et pour protéger nos concitoyens de la flambée inflationniste des prix de l’électricité.

tant pour garantir la pérennité du groupe EDF que pour faire de cette nationalisation une occasion déterminante pour améliorer les rapports, toujours complexes, entre le capital et le travail. Certes, le principe d’une détention publique intégrale du groupe est maintenu, comme la mention d’une entreprise d’intérêt national, qui laisse imaginer une protection supérieure face à tout processus de démembrement futur du groupe EDF. Néanmoins, l’abandon de dispositions importantes pour garantir l’actionnariat salarié constitue un grand défaut du texte. Nous nous étonnons que la majorité sénatoriale, que nous pensions attachée au grand principe gaulliste de la participation, ait été l’allié le plus zélé du Gouvernement pour limiter au minimum le déploiement d’un actionnariat salarié réel au sein du groupe EDF. permis, il convient de le rappeler, de garantir un partage de la valeur bénéfique pour le pouvoir d’achat des salariés, mais également de protéger davantage le groupe EDF d’un futur démantèlement boursier.

le soin d’organiser effectivement le partage de la valeur à moyen terme au sein de l’entreprise. Loin d’être anachronique, la participation constitue toujours une idée profondément moderne, alliant engagement réel des salariés dans l’entreprise, pouvoir d’achat, protection de notre souveraineté et une gouvernance plus coopérative des grands groupes.

Encore une fois, la droite sénatoriale et le Gouvernement ont choisi le conservatisme le plus obtus ; nous le regrettons. Comme notre collègue député auteur de cette proposition de loi, je ne crois pas à la bonne foi du Gouvernement quant au maintien de la propriété publique d’EDF. Comment faire confiance à un gouvernement ayant sciemment organisé le démantèlement de notre système énergétique, endetté EDF et enrichi sans raison des traders de l’énergie et l’industrie du charbon allemand ? Fidèles à notre pragmatisme et à notre soutien sans réserve à l’intérêt national, nous voterons malgré tout en faveur de ce texte, mais nous appelons le Parlement à faire preuve de la plus grande vigilance sur le futur d’EDF. En 2027, il nous faudra reconstruire notre indépendance énergétique, qu’on a laissé tomber depuis des décennies. Le défi sera grand, mais, plus que jamais, les Français attendent qu’on allège leur fardeau. Si la majorité actuelle n’a pas souhaité le faire, une majorité nouvelle le fera. Avec

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, revenons à l’hiver 2022. Nous étions quelques mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui avait engendré de vives tensions

concerne le mécanisme de fixation du prix européen, dit mécanisme de la dernière énergie appelée, la situation est tout à fait incompréhensible pour les Français, les collectivités, les entreprises et nombre d’entre nous. Nous produisons une électricité à un coût raisonnable.

et l’indemnisation des actionnaires minoritaires. L’objectif était évidemment d’empêcher tout nouveau projet de démantèlement, à l’image du funeste projet Hercule. Après le coup de rabot sénatorial, le texte actuel prévoit une contractualisation des activités du groupe EDF avec l’État et un actionnariat 100 % public.

Je centrerai mon propos sur la responsabilité de l’État, désormais détenteur de l’intégralité du capital d’EDF. L’article 2 de cette proposition de loi prévoit que, dans le cadre d’un contrat décennal, soient fixés des objectifs relatifs, entre autres sujets, à la trajectoire financière d’EDF et à la maîtrise des prix pour les ménages et les entreprises.

De surcroît, la réforme annoncée de la structure du marché européen, peu claire à ce stade, ne sera d’aucun secours sur ce point. La question est donc financière et exclusivement financière. La compétitivité du parc de production national

Nous voterons la proposition de loi de notre collègue député Phillipe Brun ; mais il revient maintenant au Gouvernement de tirer les conséquences de ce texte, en jouant le rôle qui doit être désormais le sien en tant qu’actionnaire unique et garant de l’intérêt général.

La qualification d’intérêt national de l’entreprise EDF est également essentielle, en particulier pour les enjeux de souveraineté énergétique et de transition écologique.

Mais la concrétisation de ces projets hydroélectriques dépend de l’évolution du cadre juridique et de la résolution du contentieux européen relatif au renouvellement des concessions.

En conséquence, la proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement est définitivement adoptée. ( Mes chers